La séance est reprise.

La commission pourrait accepter de modifier le fait générateur du délai de douze mois, mais la prorogation dérogatoire de six mois proposée par le Gouvernement ne peut pas être acceptée : elle viderait la mesure de son intérêt et serait, après l'adoption de la directive, contraire au droit de l'Union européenne. C'est pourquoi

peut porter préjudice à l'exploitant, si la décision est défavorable. De plus, cet amendement est contraire au principe général du droit de recours en cassation. La jurisprudence admet, pour des raisons de bonne administration de la justice, la possibilité pour le tribunal administratif de statuer en premier et en dernier ressort, mais

ensemble. Nous saluons l'équilibre trouvé par la commission, qui a aménagé la dispense de participation du public, en maintenant la concertation préalable pour les projets initialement soumis à un débat public ou à une concertation préalable, ce qui est un moindre mal. Nous craignons malgré tout un affaiblissement de la démocratie participative et que ces dispositions ne nuisent à la bonne compréhension de la planification territoriale.

un moyen de permettre aux territoires dans leur ensemble, de mieux s'approprier les projets. Cela vaut aussi pour les collectivités, qui n'ont pas toujours les moyens de s'opposer à une implantation, dès lors que celle-ci est permise

à ces dispositions. Je le répète, dans le cas où un projet similaire serait présenté dans les dix ans qui suivent, la Commission nationale du débat public (CNDP), pourra demander une enquête préalable. Celle-ci aura lieu et sera de droit. L'idée est de dispenser d'une étude supplémentaire, qui rallongerait les délais, un projet similaire au projet global ayant d'ores et déjà été adopté, à condition, évidemment, que la Commission nationale du débat public

est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ? Afin d'accélérer le déploiement des projets d'industrie verte, l'acceptabilité locale de ces projets est cruciale. La CNDP, autorité administrative indépendante, contribue à assurer cette acceptabilité en organisant les débats publics et les concertations préalables, qui permettent l'expression des désaccords de chacun dans un cadre réglementé et la prise en compte par les industriels des enjeux locaux. Exclure les projets industriels du champ des projets soumis à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable constituerait donc une régression en matière de démocratie environnementale et diminuerait l'acceptabilité de l'implantation de sites industriels.

le non-recours systématique à une commission ou une enquête publique dans le cas où un projet similaire au projet d'ores et déjà adopté serait présenté dans les dix ans qui suivent. Nous ne souhaitons pas de concertation systématique. Évidemment, si la CNDP souhaite qu'une concertation ait lieu, elle sera de droit.

ou de concertation préalable propre dès lors qu'une consultation globale a déjà eu lieu. L'article 3 prévoit déjà plusieurs cas dans lesquels ce délai est allongé, ce qui peut poser question. Il est précisé, à l'alinéa 4, que, lorsqu'un débat global ou une concertation globale a eu lieu sur un ensemble de projets, ces projets sont dispensés d'une nouvelle consultation propre, si leur mise en oeuvre démarre dans les dix ans. ce délai de dix ans nous semble beaucoup trop long. Nous pouvons entendre que, lorsque plusieurs projets similaires émergent sur un territoire homogène, un débat global puisse avoir lieu, mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence dans le temps En dix ans, beaucoup de choses peuvent changer, particulièrement à l'heure où les effets du changement climatique se font sentir et alors que les réalités d'hier ne seront pas celles de demain ... Pour nous, sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, soit les projets sur un même territoire démarrent dans les cinq ans suivant la consultation globale, auquel cas nous sommes d'accord avec la dispense de débat propre, soit ils devront faire l'objet d'un nouveau débat public propre ou d'une concertation préalable propre. L'amendement

ou le débat public et le début des travaux, qui est de sept ans. La durée de dix ans semble donc appropriée. En effet, alors que plusieurs années peuvent s'écouler entre la décision d'installation et le début des travaux, les entreprises ne disposent pas forcément d'une parfaite visibilité sur ces délais. Si le délai entre la fin du débat public

3 permet à la CNDP de se saisir, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même lorsqu'un débat global ou une concertation globale a eu lieu, de certains projets, dans le but d'organiser un débat ou une concertation, si elle l'estime nécessaire.

décisions ! La Commission nationale du débat public est très attachée à la transparence des procédures. Il semble donc nécessaire qu'elle puisse motiver sa décision. De plus, cette obligation de motivation permettrait à l'exploitant de comprendre l'origine de cette décision, et contribuerait ainsi à prévenir les conflits et les éventuels recours. En tout état de cause, puisqu'il s'agit d'une compétence discrétionnaire de la CNDP, il est probable que celle-ci motiverait sa décision même si la loi ne le prévoyait pas. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable

Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en oeuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. » L'article 3 du projet de

territoire ? Dans la situation dont il est question, un débat public ou une concertation préalable a, de fait, déjà eu lieu sur le projet. Organiser, quelques années plus tard, un nouveau débat public ou une nouvelle concertation préalable sur le même projet

n° 48 rectifié. L'accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue, citée dans le rapport Guillot sur les freins aux implantations. Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d'ouvrage, ce qui constitue autant de freins aux lancements des projets. Cet amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passé ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.

au monde économique, qui se mobilise. Nous le savons, l'accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale est attendue, car elle peut permettre la réalisation des travaux avant-

de la part des autorités administratives. Si ces délais ne sont pas tenus, les entrepreneurs pourront entamer leur projet. Il y a deux manières de voir ces amendements

Cette stabilité législative, que l'ensemble des acteurs économiques appellent de leurs voeux depuis de nombreuses années, constituerait un levier important pour la compétitivité de la France, dans un contexte de forte concurrence internationale et de crises successives.

les législations nouvelles au code de l'environnement, hors textes de transposition européenne, assurent une stabilité normative. Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d'environnement ne pourra être adopté.

des ressources doit s'accompagner d'une véritable planification sur la structuration de la filière concernée. De la formation à la gestion des déchets, les acteurs du secteur doivent être coordonnés à l'échelle des territoires et de la filière. Intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur, de la première utilisation du produit à sa fin de vie, sera déterminant pour maîtriser les risques et limiter les coûts économiques et environnementaux.

en ressources de notre industrie et de proposer une structuration adaptée des filières sur l'ensemble du cycle de vie des matières. Cela peut notamment passer par un document de planification. Mais cette intention

prévoit : « Le ministère chargé de l'écologie engagera, sur la base des travaux du comité pour les métaux stratégiques (Comes) et du premier plan national des ressources, un plan de programmation des ressources jugées les plus stratégiques en l'accompagnant d'une politique industrielle ambitieuse de valorisation du stock de matière, en particulier pour les métaux critiques contenus dans les déchets. » Dans ce cadre, dès février 2019 ont été lancés les travaux d'élaboration d'un plan de programmation des ressources minérales de la transition bas-carbone. En effet, pour construire les infrastructures énergétiques indispensables à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

un rapport sur la sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales. À cette occasion, les deux ministres avaient annoncé l'ouverture d'un appel à projets national, opéré par Bpifrance dans le cadre du plan d'investissement France 2030, et ciblé sur les métaux critiques à destination des filières industrielles. Le plan d'investissement France 2030 mobilisera ainsi une enveloppe de 1 milliard d'euros- 500 millions d'aides d'État et 500 millions de fonds propres -pour renforcer la résilience du tissu industriel sur les chaînes d'approvisionnement en métaux.

est l'économie circulaire, alors même qu'elle devrait être au coeur de notre industrie verte de demain. L'économie circulaire nous amène à nous interroger à plusieurs titres sur nos modes de production et de distribution, et d'une manière plus globale sur l'intégration d'une dimension durable dans l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de sa conception à son recyclage. Elle devrait donc être l'alpha et l'oméga de nos réflexions actuelles,

M. Fernique, qui a convaincu la commission de la pertinence de répliquer le modèle des projets alimentaires territoriaux en matière d'industrie circulaire.

soudain. La création de projets territoriaux d'industrie circulaire associant entreprises, collectivités, État et associations va dans le sens de la valorisation et de l'optimisation des ressources des territoires, au plus près de la demande. Bien sûr, le marché de ces industries dépasse souvent l'échelle du territoire, mais cet outil serait complémentaire

dite loi Agec, vient en support, mais ne répond pas au même objectif. Quant au programme Territoires d'industrie, il répond principalement aux besoins d'ingénierie au sein des territoires industriels et de soutien aux entreprises industrielles en difficulté.

madame la présidente, avant de présenter cet amendement, j'aimerais dire quelques mots sur l'article 4.

l'amendement n° 315 du Gouvernement, qui vise à simplifier la disposition relative aux résidus de production au sein des plateformes industrielles. La rédaction adoptée en commission a simplifié l'approche prévue à l'article 4. Parmi les conditions à remplir pour qu'un résidu puisse être réutilisé, le Conseil d'État avait estimé que seule était nécessaire celle qui est relative à l'absence d'incidence globale nocive. Cet amendement permet d'opérer ce recentrage en revenant à une rédaction très proche de la rédaction initiale. Je vous invite donc, monsieur le rapporteur, à soutenir

au regard du droit de l'Union européenne. La directive-cadre sur les déchets prévoit en effet que les résidus de production ont soit un statut de déchet, soit un statut de sous-produit, à condition de respecter les conditions fixées par le droit européen et le code de l'environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre, et il n'est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C'est pourtant ce que prévoit le dispositif proposé par le Gouvernement, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production issus d'une plateforme industrielle, sans pour autant faire référence à la notion de sous-produit. La commission a donc corrigé ce point afin de mieux articuler la proposition formulée par le Gouvernement avec la notion de sous-produit cadrée par la directive européenne. Je constate que le Gouvernement s'inscrit dans cette logique en amendant notre proposition, mais il le fait, à notre sens, imparfaitement puisqu'il ne retient pas l'ensemble des conditions prévues par le droit européen

La sortie du statut de déchet autorise l'incorporation des déchets dans le processus de production industrielle ; son principe est donc au coeur d'une industrie circulaire. L'absence de reconnaissance en droit français du statut de produits pour les objets exclus du statut de déchet dans les autres États de l'Union européenne pénalise notre tissu industriel. Nous sommes en effet dépendants de l'importation de nombreuses matières premières nécessaires à l'élaboration de produits manufacturés : matières premières fossiles ou minérales, mais aussi certaines matières végétales et renouvelables, introuvables en France du fait notamment de paramètres climatiques. Cet amendement vise à maintenir sur le territoire français le statut de produits pour les substances ou objets ayant fait l'objet d'une sortie du statut de déchet dans un pays de l'Union européenne.

Je rappelle que, hormis les critères pouvant être fixés à l'échelle européenne, il revient aux États membres de définir les modalités de la sortie du statut de déchet. Ces amendements visent à revenir sur ce principe en prévoyant une reconnaissance automatique par la France de la sortie du statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne. Cela reviendrait à renoncer à notre souveraineté réglementaire en la matière. Nous devrions alors adopter les mêmes normes que des pays tiers de l'Union européenne, sans que la réciproque soit assurée.

qu'une sortie du statut de déchet s'est faite à l'étranger dans les règles de l'art, ce qui permettrait une application du statut de produit aux objets ou substances concernés. Ou alors pourrait-on envisager une extension des critères communautaires de sortie du statut de déchet

soient retirés ou qu'ils ne soient pas adoptés. Nous allons continuer à travailler sur une vision européenne du déchet recyclable, car c'est l'avenir de l'industrie. Les déchets ne sont plus des déchets : ils sont en train de devenir des matières premières, mais il faut qu'ils le soient conformément aux normes de sécurité françaises.

Pour intensifier cette lutte, l'amendement que nous vous proposons vise à s'assurer que les sanctions sont appliquées, que les équipements collectés sont considérés comme des produits usagés ou comme des déchets. Les sanctions doivent en effet permettre de punir les acteurs qui alimentent les filières illégales en sortant du cadre réglementaire sécurisé, lequel garantit la conformité de traitement de ces équipements dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement

le statut de déchet s'il est utilisé dans un processus de production, quand ce résidu de production est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.

vous suivait, nous serions en contradiction avec la directive-cadre européenne relative aux déchets, qui prévoit- je vous le rappelle -que les résidus de production visés par l'amendement ont un statut soit de déchet, soit de sous-produit, à condition de respecter les conditions fixées par le droit européen et le code de l'environnement pour le statut de sous-produit. Il n'est pas possible d'inventer une troisième catégorie.

alors l'amendement pourrait conduire à desserrer très largement les exigences environnementales. En effet, il permettrait de faciliter le contournement des critères applicables à la sortie du statut de déchet. En somme, les producteurs et détenteurs de déchets pourraient réaliser des sorties de ce statut sans démarche sans démarche particulière, sinon celle de justifier du respect des conditions légales en cas de contrôle. C'était, d'une certaine manière, l'intention originelle du Gouvernement dans ce projet de loi, mais la commission n'a pas souhaité le suivre dans le suivre dans cette direction. Il ne faut pas, selon nous, ouvrir trop largement les vannes. Je rappelle que le statut de déchet a un objectif essentiel dans le code de l'environnement : celui d'éviter les risques pour l'environnement et la santé publique. Pour ces raisons

Quel gâchis !

l'utilisation de matières premières « recyclées » tout en assurant la sécurité, à la fois, des producteurs et des utilisateurs.

de renforcer la traçabilité des déchets non dangereux en l'alignant sur celle qui s'applique déjà aux déchets dangereux la mise en place de Trackdéchets. Le renforcement de la transparence des données de gestion des déchets non dangereux permet à la fois d'améliorer la lutte contre les exports illégaux de déchets et de répondre aux objectifs nationaux de développement de l'économie circulaire.

territoire ? Je partage totalement les objectifs des auteurs de ces amendements identiques n 72 rectifié et 228 rectifié : améliorer la lutte contre les exports illégaux de déchets et répondre aux objectifs nationaux de développement de l'économie circulaire. Le dispositif proposé, qui consiste à renforcer la traçabilité des déchets non dangereux, me semble répondre à ces objectifs. Je m'interroge toutefois sur la proportionnalité de cette proposition et sur son applicabilité. L'administration sera-t-elle en mesure de récolter l'ensemble de ces informations et de les traiter ? La charge sur les gestionnaires de déchets n'est-elle pas disproportionnée par rapport aux avantages induits ?

territoire ? Le règlement européen du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, fondé sur les principes de la convention de Bâle, vise à renforcer la maîtrise de cette pratique afin de s'assurer qu'un déchet faisant l'objet d'un transfert soit traité dans des conditions qui garantissent le contrôle des conséquences sur l'environnement. à encadrer différents cas de transfert, d'exportation et d'importation, et d'établissement des procédures et des régimes de contrôle en fonction de l'origine et de la destination du type de déchet transféré et du type de traitement réalisé. L'amendement proposé relève donc donc d'un champ de compétence de l'Union européenne. C'est pourquoi je me vois contraint de donner un avis défavorable.

Si un transfert illicite est constaté, une amende doit être appliquée, quel que soit le délai avec lequel le ministère est en mesure de l'infliger. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'alinéa 29. Si cet amendement venait à être rejeté, pourriez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, ce qui se passerait à l'avenir si le ministre concerné n'était pas en mesure d'appliquer une sanction dans les trois ans ? Les responsables du transfert illicite s'en sortiraient-ils sans

de ne pas limiter le délai de prescription et d'appliquer, le cas échéant, le délai de prescription légale par défaut.

en matière de réduction des coûts et, bien entendu, de lutte contre le gaspillage de nos ressources, qui se raréfient et qui- je le crains -continueront à se raréfier. Toutefois, les dérogations précises prévues à cet article doivent être bien encadrées pour ne pas ouvrir la porte à diverses fraudes la part d'entreprises cherchant à ne plus payer de taxes pour le traitement de leurs déchets sans pour autant réemployer ces derniers en tant que matière première. C'est ce qui est prévu. Aussi, nous ne comprenons pas pourquoi l'État n'aurait que trois ans pour sanctionner un contrevenant. Une fois les constatations réalisées, les investigations, la matérialisation des preuves

Nous avons en effet considéré que, en matière de transferts transfrontaliers de déchets, les procédures peuvent parfois nécessiter de longs travaux d'investigation, qui plus est avec des autorités étrangères. La suppression de toute forme de délai, comme le proposent les auteurs de ces amendements, semble toutefois excessive. Il est en effet habituel de définir une échéance au-delà de laquelle il n'est plus possible de poursuivre une personne. C'est pourquoi je donnerai un avis défavorable sur les amendements identiques n 82 rectifié, 193 et 249.

Je constate que certains se rallient aux peines plancher ... Cela pose d'évidents problèmes de proportionnalité et de légalité de la peine encourue.

de traitement des déchets concernés ». Bien évidemment, je me félicite du fait que la commission ait adopté l'amendement que j'avais proposé. Toutefois, comme il est précisé dans l'étude d'impact du projet de loi, « l'origine des trafics illicites reste l'appât du gain, soit par les économies sur le coût du traitement qu'il peut générer, soit par les bénéfices qui peuvent être issus du déchet lui-même ». En conséquence, et considérant que les opérateurs économiques procédant à de telles pratiques disposent parfois de moyens financiers importants, le dispositif retenu dans la loi doit être particulièrement dissuasif. Ainsi, le présent amendement tend à porter à dix fois le coût du traitement des déchets concernés le montant maximal de l'amende pouvant être infligée. Nous parlons bien ici d'un montant maximal : rien n'obligera à ce que ce soit systématique.

dans les chaînes de valeur de l'industrie peut réduire les émissions de CO2 de 58 % pour l'acier et de 92 % pour l'aluminium par rapport aux matières premières extraites. Il s'agit donc d'un levier majeur pour accélérer la décarbonation de l'industrie en France et notamment des filières qui sont les plus émettrices de gaz

à notre sens. Le pouvoir réglementaire dispose de la faculté d'imposer l'intégration de matières recyclées dans certains produits et matériaux. Ces obligations d'incorporation de matières recyclées pourraient au demeurant être renforcées au niveau européen. C'est pourquoi nous donnons un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Cet

Sur le fond, l'amendement était plus spécifiquement lié au fait que le développement du commerce en ligne entraînait davantage de retours et d'invendus par rapport aux canaux traditionnels de la distribution, tout particulièrement dans le domaine du textile, ce que montrent plusieurs études. Ma collègue signalait que la plupart de ces textiles invendus et retournés à leurs distributeurs n'étaient n'étaient pas remis en vente, mais exportés pour être détruits et la plupart du temps brûlés. Notre amendement vise donc à interdire la destruction ou l'exportation pour destruction des marchandises neuves du secteur de l'habillement et du prêt-à-porter.

Or force est de constater que la situation n'a pas vraiment évolué dans le bon sens. Malgré les obligations de la loi Agec dans l'incitation au réemploi et aux dons à des associations de lutte contre la précarité, une partie des invendus est toujours détruite.

toute la prudence et l'humilité dont je fais désormais preuve dans la lecture des codes, je veux dire que cet amendement nous semble satisfait par l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement créé par l'article 35 de la loi Agec. Depuis le 1 janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler les produits non alimentaires invendus qui étaient couverts par une filière à responsabilité élargie du producteur avant le vote de la loi Agec. Les produits textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison neufs sont donc concernés par cette interdiction de destruction

-interdit l'élimination des invendus de produits textiles depuis le 1 janvier 2022, que cette élimination soit effectuée en France ou à l'étranger. Je demande donc le retrait ; à défaut,

En accord avec la commission et le Gouvernement, je propose que nous poursuivions nos débats jusqu'à la fin de l'examen du chapitre IV. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre, cet amendement, élaboré en lien avec France urbaine et l'Institut national de l'économie circulaire

des friches potentiellement mobilisables. Chaque territoire de planification, à l'échelle communale ou intercommunale, doit désormais démontrer qu'il a cherché à mobiliser tous les potentiels fonciers déjà artificialisés pour ses besoins de développement, afin de répondre aux enjeux de renaturation.

Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, les communes sont déjà tenues, quand elles ont un PLU, de tenir compte des friches existantes avant d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. La question n'est donc pas nouvelle

plus petites communes ou territoires qui n'en bénéficient pas. Sachez que nous avons missionné la Banque des territoires pour réaliser ce travail, avec un dispositif qui permettra de recenser de manière exhaustive l'ensemble du foncier disponible, de le qualifier et donc de le rendre aisément disponible aux investisseurs potentiels.

clore les procédures plus vite, faire cesser les activités plus vite, libérer les terrains plus vite, tout cela uniquement pour aller plus vite et pour répondre aux préoccupations d'un certain nombre de sénateurs, dont la sénatrice Cukierman, sur la libération des friches, qui doit nous permettre de réindustrialiser des territoires industrialisés auparavant.

de se substituer à l'exploitant pour la mise en sécurité du site. Enfin, nous renforcerons le pouvoir des préfets pour faire cesser une activité en partie, et faciliter la dépollution et la réutilisation du site. Dans ce cadre, la commission des affaires économiques du Sénat, à l'occasion de l'examen de cet article, a tenu à apporter des précisions sur les modalités de détermination de cet usage futur. Je partage ces propositions. Je souhaite seulement m'assurer de leur sécurité juridique, ce qui justifie l'amendement n° 309. Cet amendement gouvernemental tend, en particulier, à supprimer la référence à des « évolutions en cours de documents d'urbanisme », qui ne sont pas opposables au moment de la saisine d'une collectivité sur l'usage futur envisagé,

En commission, nous avons restreint cette latitude afin d'éviter les « surprescriptions » en matière de dépollution des sols, qui peuvent décourager les industriels de s'installer sur des terrains précédemment occupés par de l'industrie si on leur demande ensuite de dépolluer complètement le site. Par défaut, ce dernier devra être remis dans un état qui permette un usage industriel. Il y va également de la compétitivité des entreprises qui souhaitent s'installer. Dans le même temps, nous avons aussi introduit la possibilité, pour le maire, de signaler au préfet que l'usage futur de la zone, tel qu'il est défini dans les documents d'urbanisme, est incompatible avec des prescriptions de dépollution qui seraient suffisantes pour un simple usage industriel. protection de l'environnement (ICPE) autorisées avant 2004. Il est en effet normal que les collectivités gardent la latitude de faire évoluer comme elles l'entendent leurs documents d'urbanisme. Si elles veulent changer l'usage de la zone, elles en ont parfaitement le droit. Les prescriptions de dépollution pourront alors être adaptées à ce nouvel usage. Compte tenu des délais d'évolution des documents d'urbanisme, qui peuvent atteindre plusieurs années, nous avons également précisé que, si une évolution des documents est en cours- par exemple si les consultations obligatoires sont en cours -, le maire peut également le signaler au préfet. Je souligne que ce dernier ne sera pas contraint de faire droit à la demande du maire si, d'aventure, le projet de modification de l'usage de la zone est encore très hypothétique : le préfet gardera, comme aujourd'hui, un pouvoir d'appréciation. Nous choisissons de faire confiance au bon sens du préfet,

pour les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1 juin 2022, tout en limitant le risque d'effets d'aubaine. Cependant, le projet de loi ayant été présenté au printemps 2023 étant donné qu'il ne sera pas adopté avant cet été, il est proposé d'intégrer une année supplémentaire dans cette disposition « voiture-balai » afin de rendre davantage de sites éligibles aux dispositions du présent article. Quel est l'avis de la commission ? Depuis le 1 juin

Le 3° de l'article 5 confie au préfet un pouvoir supplémentaire de mise en demeure pour faire procéder à la cessation d'activité d'une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine au motif qu'elle ne serait plus exploitée depuis trois ans, dans le but de libérer du foncier pour un usage industriel. Cette restriction au droit de propriété, garanti par la Constitution, et aux droits et à la gestion de l'exploitant se justifie par son objectif d'intérêt général, à savoir faciliter les implantations d'activités industrielles.

notamment, de libérer de tels terrains industriels pour, par exemple, étendre une surface commerciale, ou même des installations de services. Par ailleurs, le recours au décret en Conseil d'État ne me semble pas nécessaire, car il n'y a pas atteinte au droit de propriété : il s'agit non pas de saisir le terrain ni d'obliger le propriétaire à vendre, mais simplement de s'assurer qu'un industriel

qui tend à anticiper la substitution d'un exploitant par un tiers demandeur dès la notification de cessation des activités. Autrement dit, j'ai l'impression que l'on va là un peu plus loin et que l'on enfreint le droit de propriété autoriserait un tiers demandeur à interrompre l'activité d'un exploitant alors que lui-même n'a pas souhaité le faire. Nous souhaitons, évidemment, qu'un tiers demandeur puisse intervenir dès que possible pour sécuriser le site, mais après l'arrêt de l'activité. Tel est l'objet de cet amendement.

pour le tiers demandeur d'intervenir en amont de la cessation d'activité. Or c'est bien une loi d'accélération que l'on souhaite mettre en place. Il s'agit donc d'accélérer davantage la procédure par anticipation.

introduit en commission, qui est d'accélérer plus en amont encore pour faciliter la réindustrialisation. Je comprends votre argument selon lequel le préfet pourrait avoir des difficultés à se prononcer très en amont sur la viabilité du projet futur, ne sachant pas, par exemple, comment la pollution du site évoluera entre l'autorisation donnée au tiers demandeur et sa prise en charge effective du site. Mais je rappelle que c'est le préfet qui se prononce, et et qu'il conserve une marge d'appréciation sur la viabilité du projet présenté par le tiers demandeur. Il lui est loisible de refuser l'autorisation s'il estime que le projet est trop incertain. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il fait aujourd'hui ! Je rappelle également que les garanties financières peuvent être revues en cas de modification des mesures prévues initialement dans le mémoire de réhabilitation du tiers demandeur. L'administration demeurera donc libre de refuser des demandes trop en amont si leur réalisation lui semble incertaine. Il paraît complètement contre-productif de bloquer par principe l'anticipation à trois mois alors que les opérations de dépollution peuvent prendre des années ! La commission a donc émis un avis défavorable.

l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu, le cas échéant, à sa remise en état. Il peut la confier à un tiers demandeur. Mais pour le cas où le tiers demandeur serait lui aussi défaillant, il nous paraît opportun que la responsabilité de la remise en état incombe au dernier exploitant.

le préfet au tiers demandeur de prendre en charge un site est conditionnée à l'obligation de constituer des garanties financières, justement pour pouvoir mener à bien la réhabilitation prévue, même en cas de défaillance du tiers demandeur. Ces défaillances sont par ailleurs, en toute hypothèse, rarissimes puisque les tiers demandeurs s'engagent sur des projets rentables. En revanche, la perspective pour le dernier exploitant de pouvoir être « rattrapé » et de devoir se charger de la réhabilitation du site, alors même que cette responsabilité a été contractuellement transférée à un tiers, constitue un frein important pour les exploitants à s'engager dans une procédure de tiers demandeur.

face à cet enjeu et à ce défi de la requalification des friches. Nous l'avons rappelé, les friches amènent bien souvent d'autres friches.

Votre amendement vise un aspect essentiel de la mobilisation du foncier à des fins industrielles qui n'est de fait pas abordé par le projet de loi, à savoir la gestion des anciennes friches. En effet, souvent, l'exploitant a disparu.

à savoir le rachat des espaces fonciers pour aider les industriels à financer leur modernisation, ce qui reviendrait à soutenir des modes de production plus responsables de l'environnement. Nous savons par expérience l'importance pour les EPCI, qui ont désormais désormais la compétence économique, d'avoir des terrains disponibles à proposer aux investisseurs. Or les élus locaux n'ont pas toujours les leviers suffisants pour aider à l'installation ou à la modernisation des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette question puisse être étudiée à travers un rapport qui étudierait l'opportunité d'un financement de la rénovation et de la modernisation des industries par le rachat du foncier par les établissements publics de coopération intercommunale ou par des sociétés d'économie mixte communales ou intercommunales, bien sûr avec l'aide de l'État.

raison, des réflexions sont en cours dans les collectivités sur l'opportunité de constituer des foncières économiques de ce type. Cela peut être une bonne manière d'optimiser, sur un territoire, la gestion du foncier économique, et notamment industriel.

en cas d'exploitation illégale d'un site, qu'il soit ou non ICPE, de prononcer, en plus de la mise en demeure, des éventuelles mesures conservatoires et d'astreinte journalière déjà prévues, une amende dont le montant est plafonné à 15 000 euros. l'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte, notamment, de l'importance de la dégradation de l'environnement. Nous vous proposons de

un acte politique fort en créant la créance envers la planète pour les entreprises. Il s'agira d'une créance privilégiée qui va passer- c'est vous dire si Bercy lui donne de l'importance ! -avant même les créances fiscales. Nous sanctionnons ceux qui ne respectent pas les règles,

Le montant de 15 000 euros a été fixé par parallélisme avec celui qui est fixé à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour les manquements des entreprises à leurs obligations au titre du code de l'environnement. Il nous a été présenté par l'administration comme suffisant, dans la mesure où les exploitations illégales sont souvent, par nature, de petites exploitations, mais nous n'avons aucune objection à relever le plafond, dans la mesure où le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. Aussi, nous émettons un avis de sagesse sur ces deux amendements.

L'administration nous assure que ce souhait est déjà satisfait par les dispositions du code de l'environnement, et que c'est bien dans ce sens que doivent s'entendre les dispositions du du 2° du II de l'article 122-3.

Il nous apparaît important de nous assurer de la continuité de la compensation dans le passage des sites naturels de compensation aux sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR). L'amendement

que ces deux amendements

la restauration écologique peut être définie comme une action mise en oeuvre sur un milieu dégradé pour faire évoluer le milieu vers un état plus favorable à son fonctionnement ou à sa biodiversité. La renaturation se définit quant à elle comme un ensemble d'actions d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un seul non artificialisé. C'est ainsi une forme incomplète de restauration ne portant que sur le sol.

qui ont été créés récemment, la suppression de ce dispositif au profit de sites naturels de restauration et de renaturation nous laisse sceptiques. En quoi l'alternative proposée avec ces SNRR répond-elle aux complexités évoquées par les porteurs de projet, qui sont très rares, avec les sites Le nouveau dispositif est fondé sur la simple hypothèse d'un gain attendu, mais qui n'est pas nécessairement écologiquement équivalent à l'environnement détruit. En d'autres termes, ce texte maintient une simple obligation de moyens pour ces sites. Cette mesure n'est pas raisonnable. Si l'on veut garantir des compensations écologiques suffisantes et efficaces, on ne peut se limiter à une simple hypothèse. Nous proposons donc de maintenir l'obligation de résultat, telle qu'elle est prévue dans le droit en vigueur. Nous demandons enfin que les actions de compensation

risquerait de concurrencer des mécanismes déjà existants et insuffisamment mis en application par les personnes publiques. Nous pensons ici au financement des actions de restauration prévues par les documents d'objectifs Natura 2000 ou dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes sur l'eau et les milieux marins. Concentrons-nous sur l'existant plutôt

amendements ? L'article 7 prévoit de fonder l'agrément des sites naturels de restauration et de renaturation sur le gain écologique attendu par les travaux de renaturation-restauration, et non sur le gain précisément obtenu, comme dans le dispositif actuel. Ce changement découle d'un constat : le régime juridique des sites naturels de compensation a, à ce jour, été très peu appliqué. Une des raisons avancées est que la démarche d'agrément est perçue comme complexe techniquement, en particulier parce qu'elle nécessite à l'heure actuelle de préciser les gains écologiques théoriques qui seront obtenus à l'issue des opérations de restauration, alors même qu'elles ne sont pas engagées. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement, qui revient sur un apport du projet de loi susceptible de rendre plus facile l'utilisation de ce dispositif.

puissent être utilisés au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, dans le respect des principes fixés au I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement. Or, parmi ces grands principes, on retrouve l'obligation de résultat. Quand ils seront utilisés pour compenser des atteintes à la biodiversité, les SNRR auront donc une obligation d'atteindre le gain écologique visé lors de leur conception.

contribueront à l'équilibre financier des modèles économiques développés dans le cadre de ces sites. À cet égard, il nous semble donc intéressant de permettre aux SNRR de bénéficier du label bas-carbone au titre de la compensation carbone. C'est pourquoi nous donnons un avis favorable sur l'amendement

auteurs. L'avis est défavorable. Enfin, l'article L. 163-1 du code de l'environnement porte sur la compensation des atteintes à la biodiversité, et non pas sur la compensation des émissions de carbone. Ce sont deux sujets distincts, même s'il peut exister des synergies entre l'un et l'autre. C'est pourquoi nous donnons un avis défavorable

le compte de M. Gillé. Il vise à rappeler le rôle important qu'occupent actuellement les départements dans le cadre de leurs compétences concernant les espaces naturels sensibles. Ceux-ci visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels par la mise en place de politiques de protection, de gestion et d'ouverture au public. Ils s'inscrivent donc dans une logique durable et partagée des espaces naturels. L'article 7 du présent projet de loi tend à créer, dans le cadre de la compensation environnementale, des sites clés en main dénommés sites naturels de restauration et de renaturation. L'objectif de cet amendement est de rappeler

qui pourraient être mis en oeuvre sur leur territoire. Cela permettrait certainement de coordonner les politiques publiques au niveau départemental. Pour autant, faut-il confier aux départements un rôle d'évaluation de la qualité environnementale des SNRR, alors même qu'ils ne sont pas

le plan national santé environnement et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Il s'agit de donner du crédit aux activités régénératrices qui respectent ce principe. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement territoire ? Le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement constitue un principe essentiel du droit de l'environnement, qu'il ne faut modifier

Plutôt que d'éviter ou de réduire, il est toujours plus simple de compenser en plantant des arbres ici ou là ou en défrichant un espace qui sera, plus tard, utilisé par un autre porteur, lequel compensera à son tour, et ainsi de suite Ce projet de loi porte d'ailleurs l'ambition de proposer des compensations clefs en main en son article 7, dont nous venons de débattre. Par cet amendement, nous proposons d'être un peu plus regardants sur les projets qui auraient une incidence environnementale forte

cette proposition d'implantation alternative sera présentée, pourra ainsi démontrer toute sa volonté de participer au verdissement de nos aménagements et de notre industrie, conformément à l'intitulé du projet de loi.

Le I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement précise par ailleurs, que, si les atteintes liées à un projet « ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. » Cet amendement me semble pleinement satisfait par le droit en vigueur

de cette ressource essentielle doit être considérée par l'industrie non pas comme une contrainte, mais bien comme un atout. Le présent amendement tend à ce que les entreprises qui bénéficieront des dispositifs et des soutiens financiers prévus dans ce projet de loi et, plus globalement, dans la stratégie Industrie verte, puissent rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l'impact de leurs projets industriels sur la biodiversité. Il traduit, en ce sens, le point 38 de l'avis du Conseil

de la stratégie Industrie verte. Depuis plusieurs années, les sénateurs de mon groupe militent pour l'application d'un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public. Lors de l'examen de chaque projet de loi de finances, nous faisons des propositions dans ce sens,

bénéficieront des dispositifs et des soutiens financiers prévus dans ce projet de loi et, plus globalement, dans la stratégie Industrie verte, puissent rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l'impact de leurs projets industriels sur la biodiversité.

de l'aménagement du territoire ? Nous partageons l'intention des auteurs d'assurer une reddition des comptes de la part des entreprises bénéficiant des dispositifs créés par le projet de loi Industrie verte ou par la stratégie de réindustrialisation verte du pays.

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 96 amendements au cours de la journée. Il en reste 139 à examiner sur ce texte.